sémantique ne s'accompagnait initialement d'aucune autre évolution, puisque seules les autorités organisatrices de transport proposant déjà des transports collectifs pouvaient instituer le nouveau versement, avec des contours identiques

de financements nouveaux, cet élargissement des compétences aux mobilités dites actives ou partagées pourra se traduire par une baisse du financement des transports collectifs, ce qui n'est pas acceptable. Aussi avons-nous proposé un certain nombre de financements nouveaux. Là où le transport collectif existe déjà, nous proposons de rehausser les plafonds et d'instaurer le versement mobilité dès le premier salarié, une proposition malheureusement déclarée irrecevable. Pour l'Île-de-France, dont la spécificité n'est plus à démontrer, en termes tant d'infrastructures que de potentialités de financement, il est maintenant urgent d'augmenter les taux dans les territoires les plus riches, où les entreprises bénéficient de bonnes conditions de mobilité. cette évolution depuis longtemps, et l'arrivée du Grand Paris Express, avec l'accroissement de l'offre de transport, devrait la rendre plus facile. Malheureusement, là encore, notre amendement a été déclaré irrecevable. Enfin, nous proposons l'instauration au niveau régional d'un versement transport permettant de répondre aux enjeux de maintien de l'offre de TER, donc de lignes de vie, de mobilité du quotidien, comme vous aimez les appeler, madame la ministre.

article sanctuarise le versement transport, qui devient un versement mobilité, comme ressource fiscale des autorités organisatrices de la mobilité, bénéficiant à l'ensemble des compétences

Les augmentations régulières des taux, le manque de dialogue avec les employeurs sur l'utilisation du versement transport, notamment sur la prise en compte des besoins des entreprises, l'instauration de la gratuité décidée par certaines collectivités territoriales sans concertation avec les entreprises fragilisent l'acceptabilité de cet impôt. Je suis convaincue que, pour préserver cette ressource, il faut être à la fois exigeant et raisonnable. Il faut être exigeant, notamment, en matière de transparence et d'utilisation de cet impôt.

Le Gouvernement est défavorable à ces mesures, qui se traduiraient par une pression fiscale accrue sur les employeurs. Il me paraît important de maintenir un équilibre entre les différentes sources de financement des transports en France, dont les usagers et les collectivités La commission a introduit un versement mobilité réduit à 0,3 % pour les autorités organisatrices qui n'organisent pas de services de transport réguliers.

Clairement, la question des moyens est essentielle. Il est normal, bien sûr, d'être attentif à l'existence de ressources pour les collectivités

réflexion doit nécessairement s'articuler avec les réflexions en cours sur la fiscalité locale, à la suite de la suppression de la taxe d'habitation. Dans le cadre de cette réflexion sur la fiscalité locale, je serai attentive à ce qu'une réponse soit apportée

Évidemment, les entreprises qui pratiquent ce mode de travail ne doivent pas être pénalisées par le versement transport et les taxes qui alourdissent les charges des entreprises. Nous proposons donc de donner

Quel est l'avis de la commission ?

le dispositif. Le sous-amendement vise à préciser que cette exonération est accordée à concurrence de la part du volume horaire effectué à distance. C'est un complément intéressant, qui permettra de mieux lier à la part de télétravail le niveau de l'exonération du

à transporter les salariés qui ont besoin des transports en commun pour se rendre au travail. Si l'on ne se

vote. Sans remettre en cause la nécessité de pousser les entreprises vers le télétravail, je signale qu'il est rarissime qu'un salarié fasse du télétravail

six amendements faisant l'objet d'une discussion commune. L'amendement n° 140, présenté par Mme Assassi,

que c'était un véritable débat. Vous aviez indiqué, madame la ministre, que ce sujet serait au coeur des débats de la loi d'orientation sur les mobilités. Ça y est, nous y sommes ! C'est pourquoi nous déposons de nouveau cet amendement. Le budget transport est passé au fil des années au premier plan du budget général dans de nombreuses régions. Or celles-ci dépendent, pour la quasi-totalité de leurs ressources, des moyens que l'État consent à leur attribuer, lesquels ont une forte tendance à diminuer dans le cadre des politiques d'austérité poursuivies par le gouvernement actuel. L'accentuation des baisses de dotations pénalise l'ensemble des politiques publiques menées par les collectivités et, surtout, les politiques de transport. Il est impératif de garantir aux régions, dans un contexte budgétaire extrêmement tendu, de nouvelles ressources, notamment pour assurer le renouvellement du matériel ferroviaire et améliorer l'offre de transports collectifs de voyageurs. Au travers de la mise en place d'un versement transport régional, les collectivités bénéficieraient d'une ressource propre pérenne et dynamique, qui, avec les dotations de l'État et les ressources de la billettique, contribuerait à financer le fonctionnement et les investissements des transports de voyageurs d'intérêt régional, sans avoir à fermer, comme vous le préconisez, les petites lignes. Car, derrière les mots, il faut simplifier l'exercice de la compétence mobilité par les collectivités, afin que ces dernières puissent mettre en place des solutions simples et adaptées aux besoins c'est bien la rétraction du réseau ferroviaire régional qui se profile. Notre proposition va également dans le sens de la transition écologique, en donnant aux régions les moyens de mener une politique ferroviaire ambitieuse à l'échelle de leur territoire. Enfin, les estimations dont nous disposons montrent que, sur la base d'une telle taxation, la ressource potentielle s'élèverait à un peu plus de 850 millions d'euros. Tel est le sens de notre amendement.

réduit, plafonné à 0,3 %, pour les autorités organisatrices de la mobilité qui n'organisent pas de services réguliers. Pour ma part, je partage tout à fait le point de vue selon lequel des services réguliers ne sont pas indispensables pour tous les territoires et que les autorités organisatrices doivent, lorsqu'elles mettent en place d'autres types de réponses, disposer de moyens adaptés. Toutefois, le choix pour dégager des ressources conduirait à augmenter considérablement le nombre de petits établissements redevables d'un impôt dont je voudrais redire la très grande complexité à la fois en termes de calcul et de perception. D'autres solutions semblent préférables, auxquelles le Gouvernement est en train de travailler dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, rendue nécessaire par la suppression de la taxe d'habitation. Aussi, je vous propose de supprimer cette proposition de versement mobilité plafonné à 0,3 %, étant entendu que le Gouvernement sera conduit à faire des propositions prochainement.

la spécificité française est telle que les entreprises contribuent énormément à l'organisation des transports, et ce, en réalité, d'une manière anormale.

carrément la spécificité française qui compte. Aussi, j'aurais aimé que le Gouvernement nous donne d'autres pistes de réflexion plutôt que de parler d'une prochaine révision de la fiscalité. Tel est l'objet de cet amendement, qui traduit un ras-le-bol : le ras-le-bol des usagers, des entrepreneurs et de ceux qui veulent travailler sans subir de nouvelles

étant identique à celui de mon collègue Philippe Dominati, je ne répéterai pas ce qu'il a excellemment dit, ni ce que d'autres ont indiqué, notamment notre collègue Laurent Duplomb. Néanmoins, permettez-moi d'ajouter deux ou trois éléments. Dans ce même hémicycle, voilà plus d'un siècle, l'un nos éminents prédécesseurs qui siégeait juste derrière la place

alourdir la fiscalité des entreprises, notamment dans les zones périphériques ou rurales, c'est évidemment minorer, éroder leur attractivité et leur compétitivité. Pour autant, la question soulevée par Didier Mandelli, celle de l'enclavement, de l'isolement, de la mobilité dans ces zones, est bien réelle, et il faut la prendre en considération. Le problème, c'est donc le financement. Vous choisissez de financer, mon très cher collègue, par l'impôt.

les ressources fiscales qui existent et qui sont directement fléchables en ces

qui ne souhaitent pas organiser de services réguliers de transport de personnes d'instaurer un versement mobilité à taux réduit de 0,3 % pour financer des services de mobilités actives ou relatifs aux usages partagés de véhicules

prévoit, dans ses alinéas 12 et 13, que les communautés de communes qui n'organisent pas de services réguliers de transport public de personnes peuvent instaurer ce versement. Mais, tel que placé dans le texte, il leur serait également possible de bénéficier du bonus « communes touristiques », lequel permet de majorer de 0,2

traduisent avant tout les lacunes de ce texte à son arrivée, ici, au Sénat. On peut vouloir décréter la fin des zones blanches de la mobilité, mais, si l'on n'a pas de financements pour la mise en oeuvre des moyens

l'amendement n° 140, comme je l'ai indiqué, les régions n'ont pas exprimé la demande de bénéficier du versement transport. Un prélèvement additionnel entraînerait une hausse importante de la pression fiscale puisqu'il affecterait toutes les entreprises sur l'ensemble des territoires.

nous avons considéré que ce sont les territoires peu denses, les collectivités les moins dotées sur le plan économique et en termes de services publics qui ont le plus besoin de mobilité. cas-là, les distances ont une dimension beaucoup plus contraignante pour nos concitoyens. C'est pour cette raison que nous avons fait sauter le verrou du versement régulier. On ne va pas mettre des autocars et des trains

des ressources pour financer les services de mobilité, mais il faut aussi prendre en compte l'impact sur nos entreprises. Les régions n'ayant rien demandé,

des sénateurs. Notre rapporteur a bien posé le problème. Il existe des zones blanches de mobilité, auxquelles nous voulons répondre,

Demain, des communautés de communes se verront confier l'autorité organisatrice de mobilité, ex-autorité organisatrice de transport, sans moyens.

les moyens nécessaires pour permettre aux collectivités d'assumer leur rôle dans la politique de mobilité, notamment dans les territoires ruraux.

ailleurs, on le sait bien, les entreprises vont puiser, dans leur environnement, les ressources qui sont, parfois, indispensables à leur fonctionnement. Parmi ces ressources, on trouve, bien évidemment, les ressources humaines.

Si vous examinez bien la proposition qui vous est faite, mes chers collègues, nous avons effectivement mis en place un versement mobilité facultatif, laissé à l'initiative de la collectivité, à hauteur de 0,3 %, mais nous y avons adjoint un mécanisme supplémentaire-

le mot « impôt » n'est pas forcément un gros mot ; tout dépend ce que l'on en fait ! C'est comme le cholestérol, il y a le bon et le mauvais ! Exactement ! Je suis élu local de la partie la plus pauvre du département des Ardennes, qui, lui-même, est déjà un département pauvre.

couverture du territoire en termes de mobilité, soit, selon ses propres dires, de supprimer les zones blanches de la mobilité et de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'assignés à résidence. Pour ce faire, il propose de donner aux intercommunalités la compétence en matière de mobilité. Très bien

de suivre l'exemple de nos collègues Paccaud et Duplomb en retirant votre amendement ; vous enverriez alors un signal fort aux territoires. Encore une fois, on ne peut pas imposer aux communautés de communes une nouvelle compétence aussi importante et aussi onéreuse sans rien prévoir. Ce n'est pas sérieux

: La parole est à M. Olivier Léonhardt. Cet amendement concerne le versement transport. Comme je le disais déjà hier, en Île-de-France, les départements à forte densité démographique bénéficient d'un maillage fort en transports en commun pour desservir les zones d'emploi. Au regard des déséquilibres croissants entre les zones très denses et le reste de l'Île-de-France, au regard des disparités importantes en matière de dessertes ou de répartition des investissements, un effort supplémentaire doit être demandé aux entreprises du coeur de l'agglomération. Il est normal que ceux qui bénéficient de la grande majorité des infrastructures de transport soient davantage mis à contribution., dans les départements à faible densité démographique, les entreprises sont sont bien trop souvent pénalisées par le manque de dessertes et les difficultés liées à la régularité des transports en commun. Par cet amendement, je propose de majorer le versement transport de 5 % dans les départements franciliens d'une densité supérieure à 7 000 habitants au kilomètre carré et d'appliquer un abattement de 5 % dans les départements franciliens d'une densité inférieure à 2 500 habitants au kilomètre carré. En clair, la majoration concernerait Paris et les Hauts-de-Seine, qui concentrent l'essentiel des richesses régionales. En petite couronne, les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ne seraient pas concernés au regard des autres difficultés auxquelles ils sont confrontés. L'abattement de 5 % concernerait quant à lui l'ensemble des départements de la grande couronne, là où les difficultés de transport sont les plus importantes.

juste rappeler ce que subissent les entreprises qui s'installent en grande banlieue, en particulier en matière de transport.

Cette simple péréquation ne vise qu'à inciter les entreprises à s'installer en banlieue, ce qui me semble aujourd'hui un enjeu majeur.

Dans la suite des débats que nous venons d'avoir, nous souhaitons, par cet amendement, donner aux plus de trois cents autorités organisatrices de la mobilité des ressources nouvelles pour financer les besoins croissants en matière de mobilité, ainsi que les compétences nouvelles confiées par le présent projet de loi en matière de mobilité propre et partagée. Nous prenons bien sûr acte des efforts du rapporteur pour donner des ressources nouvelles limitées aux autorités organisatrices qui n'ont pas encore de transports collectifs. Nous prenons également acte, comme l'a rappelé Hervé Maurey, du principe, énoncé à l'article 2, de l'affectation d'une partie du produit de la TICPE aux collectivités dans le cadre de leur compétence en matière de mobilité. Il s'agit d'une avancée significative et d'un signe fort. Pour autant, nous considérons que les employeurs doivent aussi participer à ce bond significatif en termes de développement de l'offre de mobilité. Actuellement, la principale ressource des autorités organisatrices de transport collectif est le versement transport des entreprises, mais leur capacité d'en fixer le taux est limitée par des taux plafonds particulièrement bas, en particulier pour les petites et moyennes agglomérations, où la part modale de l'automobile est la plus importante. Le taux du versement transport a augmenté de façon importante durant les dernières années en Île-de-France, mais cela n'a pas été le cas en province. Nous préconisons ainsi de relever les plafonds des taux de versement transport, devenu versement mobilité, pour l'ensemble des autorités organisatrices qui développent déjà des offres de transport collectif. Il s'agit également de garantir, dans un cadre de ressources contraintes qui se conjugue avec la baisse des dotations, que les crédits actuels servant au financement des transports collectifs ne soient pas détournés au profit du développement d'autres offres de mobilité, notamment celles dont le support serait la route. En augmentant les plafonds, nous laissons le choix- j'insiste sur ce mot -aux collectivités de déterminer le niveau soutenable de financement des transports par les entreprises, dans des proportions qui restent très faibles. Il s'agit bien d'un outil supplémentaire que nous mettons à disposition des collectivités- et non d'une obligation -pour développer leur offre de service public de transports. Quel est l'avis de la commission ? Je regrette